Monsieur le président, monsieur le président

de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Cela a abouti à la condamnation de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, qui était gestionnaire du site. Ce régime de responsabilité se révèle donc manifestement inadapté à la pratique actuelle de nombreuses activités de plein air : escalade, trail, rafting, jeux de piste, etc. Ces activités se déroulent souvent sans supervision directe, voire sans connaissance du propriétaire ou du gestionnaire des sites. Il y a donc

les propriétaires et gestionnaires supportant une responsabilité disproportionnée par rapport à leur capacité réelle à fournir les équipements ou l'encadrement de sécurité adaptés aux sites dont ils ont la garde. dans de nombreux cas, il paraît difficilement justifiable d'engager cette responsabilité sans faute. En poussant le raisonnement, pourquoi le propriétaire serait-il responsable de la blessure

de la responsabilité en faveur des propriétaires et gestionnaires des sites, afin de leur permettre d'offrir des conditions saines de pratique des sports et activités de pleine nature. Cette idée n'est pas entièrement nouvelle. effet, l'article L. 365-1 du code de l'environnement marque déjà un infléchissement en faveur des propriétaires et gestionnaires publics de certains terrains

dans ce domaine est donc parfaitement légitime et utile. Qui plus est, il y a ici une possibilité pour le Sénat d'agir comme force de proposition et d'entamer une réflexion qui s'inscrira dans la préparation de la prochaine réforme du droit de la responsabilité civile. Mais de cette réforme, j'entends parler depuis une dizaine d'années, et c'est d'ailleurs parce qu'elle devait intervenir que l'on ne souhaitait pas modifier le code civil à la suite de la jurisprudence

Cette proposition de loi crée, par son article 1, un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité sans faute au bénéfice de tous les propriétaires et gestionnaires de sites naturels. Ce faisant, elle

que nous proposons est équilibré. Il permettra de mieux protéger les propriétaires contre la mise en cause de leur responsabilité pour des dommages sur lesquels ils n'ont que peu ou pas du tout de prise. Cette dérogation

Toujours selon cette enquête, ces activités ont un impact socio-économique non négligeable, puisque les sports et loisirs de nature généreraient près de 6 milliards d'euros de dépenses par an. La proposition de loi que nous examinons vise à favoriser le développement de ces activités qui s'exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car elles constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales. Or ce développement serait entravé par une application stricte du droit commun de la responsabilité civile. En effet, ces espaces sont soumis au régime de la responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil,

le propriétaire d'un site naturel- ou son gestionnaire s'il avait transféré à celui-ci sa garde juridique par convention -peut voir sa responsabilité civile engagée pour des branches qui tombent ou des pierres qui roulent, dès lors que la victime démontre que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, alors même que le gardien n'a commis aucune faute. Il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité, sauf à prouver l'existence d'un cas de force majeure- force majeure- notion appréciée très strictement par les juges -ou d'une faute de la victime. L'article unique de la proposition de loi prévoyait donc de compléter l'article L. 365-1 du code de l'environnement, pour basculer d'un régime de responsabilité du fait des choses vers un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel. Bien que partageant l'objectif des auteurs de la proposition de loi, la commission a estimé que ce texte suscitait certaines interrogations, auxquelles il était nécessaire d'apporter des réponses précises. Une première interrogation sur l'opportunité même d'une intervention du législateur. Le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires du fait de dommages causés sur des sites naturels est peu abondant, voire inexistant, ces dernières années pour les personnes publiques.

C'est la première question que j'ai posée en ma qualité de rapporteur. La commission a estimé que la quasi-absence de contentieux en matière de responsabilité civile des gestionnaires et propriétaires de sites naturels n'est pas un argument en faveur du. Elle est surtout révélatrice de la très grande attention portée, nous nous dit-on, par les fédérations, en particulier à la sécurité des pratiquants de sports de nature. La commission a donc considéré que l'important développement de ces pratiques de plein air justifiait pleinement d'anticiper les difficultés à venir et les éventuels tâtonnements jurisprudentiels par par la fixation de règles précises. Fallait-il ensuite s'opposer à la création d'un nouveau régime spécial, alors même qu'une grande réforme de la responsabilité civile est annoncée par la Chancellerie ? Le président Retailleau l'a dit, les réticences qui ont été exprimées sont parfaitement compréhensibles. Cependant, il me semble utile de rappeler que, faute d'évolutions législatives depuis 1804, la responsabilité du fait des choses est devenue une construction jurisprudentielle, engagée à la fin du XIX siècle pour prendre en considération des problématiques qui n'existaient pas lors de l'élaboration du code civil. Comme il l'a déjà fait pour certaines situations spécifiques, le législateur est donc, à notre avis, tout à fait légitime à intervenir pour créer un régime adapté aux contraintes particulières inhérentes à ces sites naturels. Fallait-il alors attendre le grand projet de réforme de la responsabilité civile annoncé par le ministère de la justice pour intervenir ? La commission des lois a

S'agissant du dispositif de la proposition de loi lui-même, la commission a considéré qu'il soulevait des difficultés d'articulation avec le reste de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, d'une part, et des difficultés d'application en raison de l'imprécision des notions utilisées, d'autre part. À titre d'exemple, l'utilisation de la notion de « responsabilité civile » posait question. Si elle couvrait, certes, la responsabilité délictuelle, elle englobait également la responsabilité contractuelle du propriétaire ou du gestionnaire, ce qui n'était pas, je pense, l'objectif des auteurs du texte. Le dispositif aurait permis une exonération totale de responsabilité de ces personnes, hors les cas où elles ont commis une faute. Ainsi, un manquement non fautif à l'obligation de sécurité mise par la jurisprudence à la charge de l'exploitant d'un site payant n'aurait plus permis d'engager la responsabilité de cet exploitant à l'égard de la victime du dommage. Il en aurait résulté un transfert du risque pesant actuellement sur l'exploitant, d'une station de ski souvent professionnel et bien assuré, vers son client, seulement couvert- et encore, ce n'est pas toujours le cas -par une assurance de dommages personnels. Autant dire qu'il n'était pas possible d'en rester à la notion de responsabilité civile simple. Il fallait scinder très clairement les notions de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle. Quant au champ des personnes bénéficiaires de cette exonération, la référence aux « propriétaires et gestionnaires de sites » ne permettait pas de couvrir l'ensemble des gardiens potentiels de la chose. potentiels de la chose. du locataire si l'on ne vise dans la loi que le propriétaire ou le gestionnaire du site ? Enfin, l'utilisation de la notion de « circulation du public » était également problématique, car elle pouvait renvoyer à la circulation d'engins motorisés

La rédaction retenue écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens des sites dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. Puisque le régime de responsabilité de plein droit ne pourrait plus s'appliquer, la responsabilité du gardien du site dans lequel a eu lieu le dommage devrait être recherchée sur le fondement de la faute, comme le souhaitent les auteurs du texte. Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques, bien connue dans le domaine sportif, en vertu de laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences, ce qui revient à alléger ou supprimer la responsabilité de l'auteur ou du responsable du dommage. Cette théorie a été progressivement délaissée par la jurisprudence pour faire bénéficier les victimes du régime plus favorable de la responsabilité de plein droit du fait des choses. Le développement des assurances dans le domaine du sport n'a sans doute pas été étranger à cette évolution. En restaurant ladite théorie, la commission vous propose de revenir, dans le domaine des sports de nature et des activités de loisirs, à une conception plus limitée de la responsabilité sans faute, qui a seulement pour objet de protéger la victime contre des risques créés par autrui, et non contre des risques auxquels elle participe volontairement par son activité. Il en résulte une solution équilibrée de partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gestionnaire du terrain, qui doit mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer des conditions de sécurité optimales à l'exercice des sports et des activités de loisirs de nature, et les pratiquants, à la recherche d'une nature intacte, qui doivent prendre conscience que, malgré toutes les diligences entreprises par le propriétaire ou le gestionnaire du site- le gardien -, le « risque zéro » n'existe pas quand on pratique l'escalade, l'alpinisme, le vélo ou la randonnée dans des sites naturels peu ou pas aménagés. La commission a ensuite choisi d'introduire ce dispositif dans le code du sport, au sein des dispositions relatives aux sports de nature, plutôt que dans le code de l'environnement, puisqu'il concerne la pratique de ces sports et les activités de loisirs de plein air qui s'en approchent. La commission a estimé enfin que, puisque le jeu de la responsabilité du fait des choses était désormais écarté, les indications données au juge pour apprécier cette responsabilité, prévues à l'article L. 365-1 du code de l'environnement, n'avaient plus lieu d'être.

la proposition de loi qui vient aujourd'hui en discussion a pour objectif, en modifiant le régime de responsabilité auquel sont soumis les gardiens de sites naturels ouverts au public, d'encourager le développement des sports de nature, qui, comme cela a été rappelé, constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales. Le Gouvernement ne peut que souscrire à un tel objectif, auquel vous me permettrez d'ajouter, plus largement, celui de favoriser la plus large ouverture au public, y compris aux simples promeneurs, des espaces naturels de notre pays, dans des conditions compatibles avec les nécessités de leur conservation. Les préoccupations des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels, qui ne doivent pas être dissuadés d'ouvrir ces espaces au public en raison d'un risque excessif de mise en cause de leur responsabilité, sont à cet égard légitimes. Si la Si la proposition de loi suscite des réserves, c'est donc non pas en raison des objectifs qu'elle poursuit et des préoccupations auxquelles elle entend répondre, mais plutôt des moyens qu'elle emploie. emploie. En l'état actuel du droit, une adaptation du régime de responsabilité des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels est déjà prévue à l'article L. 365-1 du code de l'environnement. Cette disposition a été introduite en 2006 à l'occasion du vote d'une loi relative aux parcs nationaux et parcs naturels. Elle ne modifie pas le régime de responsabilité applicable, mais, en cas d'accident, elle invite le juge à apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de certains espaces naturels, en tenant compte des caractéristiques particulières de ces espaces, qui, pour des raisons de conservation des milieux, ne peuvent faire l'objet que d'aménagements limités. proposition de loi va plus loin : dans sa version issue des débats en commission, elle prévoit, au nom de la théorie de l'acceptation des risques, de substituer au régime de responsabilité actuellement applicable devant le juge civil, qui est le régime de responsabilité objective du fait des choses, un régime de responsabilité pour faute, inscrit désormais non plus dans le code de l'environnement, mais dans le code du sport. une telle évolution nous paraît prématurée, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, il serait excessif de décrire l'état du droit actuel comme permettant l'engagement automatique de la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels en cas d'accident. Certes, le régime de « responsabilité du fait des choses » que les juridictions civiles appliquent aux propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels est un régime de responsabilité sans faute. les juridictions, lorsqu'elles sont saisies d'actions en responsabilité, procèdent à une appréciation circonstanciée des faits de l'espèce. Elles recherchent notamment la réalité du rôle causal de la chose et tiennent compte du comportement de la victime pour, le cas échéant, exonérer le gardien de sa responsabilité ou atténuer celle-ci. À cet égard, comme cela a été rappelé lors des travaux en commission, il faut relativiser la portée du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse de 2016- commission des lois et M. le rapporteur y ont fait référence -, mentionné dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, qui a condamné la Fédération française de la montagne et de l'escalade, en sa qualité de gestionnaire d'une falaise, à indemniser les victimes d'un accident d'escalade.

très faible, alors que, pour ne citer que les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites du Conservatoire du littoral, la fréquentation cumulée est de 54 millions de visiteurs par an.

je rappelle que, comme votre commission en est parfaitement consciente, le ministère de la justice travaille actuellement à un vaste projet de réforme de la responsabilité civile.

Ce projet sera l'occasion de faire évoluer certains régimes de responsabilité particuliers- je suis certaine que vous y travaillerez de concert avec nous, puisque ce sujet vous tient à coeur

l'abandon par la Cour de cassation de la théorie de l'acceptation des risques en matière sportive, pour écarter l'application du régime de responsabilité du fait des choses dans certains cas de dommages matériels causés par un pratiquant sportif à un autre pratiquant. Dans ce contexte, introduire aujourd'hui dans le droit positif une nouvelle disposition dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile paraît prématuré. cru comprendre, au travers de vos débats en commission, que nombre d'entre vous n'étaient pas insensibles à la nécessité d'une réflexion élargie à l'ensemble du droit de la responsabilité civile. troisième raison qui motive notre avis : la rédaction de la proposition de loi issue des travaux en commission, si elle résout certaines difficultés soulevées par la rédaction initiale du texte, paraît problématique à d'autres égards. Ainsi, cette rédaction ne fait pas référence à la responsabilité administrative, au contraire de l'actuel article L. 365-1 du code de l'environnement, qui invite également le juge administratif, le litige relève de sa compétence, à tenir compte des contraintes tenant aux nécessités de la préservation des espaces naturels. Cela pourrait conduire à des conditions d'indemnisation différentes selon le juge compétent, alors que, en l'état, dans des cadres théoriques certes distincts, le juge judiciaire et le juge administratif parviennent généralement à des résultats très similaires.

Il semble en effet nécessaire de limiter expressément ce champ d'application aux seuls espaces « naturels », dès lors que les activités de loisirs peuvent également être pratiquées en dehors de tels espaces, notamment en milieu urbain. Enfin, et surtout, Enfin, et surtout, votre commission propose, en contrepartie de la création d'un nouvel article dans le code du sport, d'abroger purement et simplement l'article L. 365-1 du code de l'environnement. Or le nouveau dispositif ne couvre pas la totalité des champs traités par cet article : en particulier, il ne traite pas de la circulation des piétons. Ce faisant, la proposition de loi laisse sans réponse les préoccupations, à cet égard, des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels, lesquelles sont pourtant au coeur de votre travail. Cette difficulté ne saurait d'ailleurs se régler par un simple élargissement du champ d'application du texte de la commission si l'on peut trouver légitime d'opposer l'acceptation du risque à un sportif qui pratique en toute connaissance de cause une activité risquée, il en va différemment en ce qui concerne le simple promeneur, et le Gouvernement ne saurait souscrire à un texte qui conduirait à un affaiblissement du droit des victimes. À cet

Dans ces conditions, le Gouvernement pourrait souscrire à un texte qui, sans modifier le régime de responsabilité applicable, viendrait étendre le champ d'application, actuellement trop restrictif, de l'article L. 365-1 du code de l'environnement, initialement visé par la proposition de loi. C'est pourquoi vous est soumise par voie d'amendement une proposition de réécriture de cet article, afin d'élargir son champ d'application à l'ensemble des personnes propriétaires ou gestionnaires, ainsi qu'à l'ensemble des « espaces naturels ». La liste La liste des personnes publiques dressée par l'actuel dispositif, qui ne mentionne que l'État et la commune, est en effet trop restrictive. Celle des espaces concernés l'est également, puisque seuls sont visés certains espaces particulièrement protégés. C'est C'est ainsi que, dans le cas jugé par le tribunal de grande instance de Toulouse, l'article L. 365-1 du code de l'environnement ne pouvait trouver à s'appliquer, le lieu de l'accident ne figurant pas sur cette liste.

je l'ai indiqué, c'est une réflexion qui aura toute sa place dans le cadre de la réforme globale du droit de la responsabilité civile qui a été engagée par le Gouvernement. en l'état, il importe, tout en adaptant son champ d'application, de conserver l'économie générale d'un dispositif qui permet de concilier le droit commun de la responsabilité tant civile qu'administrative et la la prise en compte des contraintes spécifiques des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels, tout en garantissant une protection satisfaisante du droit des victimes. La parole est à M. Loïc Hervé, pour

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la période contemporaine est marquée par un attrait croissant pour les sports et activités de pleine nature. Il faut se féliciter de ce phénomène, qui favorise le développement touristique, donc économique, de nos territoires et valorise des espaces naturels. Le département dont je suis l'élu, la Haute-Savoie, est particulièrement concerné par ce phénomène. Je ne vais pas vous citer ici l'ensemble des activités extérieures qui sont pratiquées chez nous tout au long de l'année, mais simplement vous rappeler quelques disciplines montagnardes emblématiques comme l'escalade, l'alpinisme, le ski, le parapente et, plus récemment, le trail. Ces activités, comme la plupart des activités de nature, sont par essence à risque, et les pratiquants de ces sports le savent. Ce constat doit nous amener à remarquer une forme de paradoxe

Le texte que nous proposent aujourd'hui nos collègues a suscité une double réaction au sein de notre groupe. Première réaction, partagée par les précédents orateurs : orateurs : appliquer de manière brutale la responsabilité du fait des choses au propriétaire ou au gestionnaire de sites pour des dommages causés lors d'une pratique sportive sur des sites naturels pose problème. En effet, cela va provoquer un découragement, donc probablement un désengagement, des fédérations sportives, voire des collectivités qui s'étaient organisées pour accompagner et développer ces activités. On comprend alors aisément les répercussions immédiates en matière d'attractivité touristique que cela pourrait engendrer dans nombre de territoires. Deuxième réaction : le problème de droit

Se pose alors une question de principe : peut-on, doit-on, légiférer maintenant ? Au-delà du fait que ce soit une décision judiciaire isolée, on pourrait aussi se dire qu'il serait préférable d'attendre les travaux de notre Haute Assemblée sur le projet de de réforme du droit de la responsabilité qui devrait s'amorcer à la fin de l'année. Mais, là encore, est-ce une raison pour nous empêcher de travailler dès maintenant ? Non ! Notre présence en nombre ce soir montre combien cette question nous Après une réflexion alimentée par les travaux approfondis de notre rapporteur et de la commission des lois, nous avons estimé qu'il était nécessaire que le Sénat s'attaque, dès aujourd'hui, au problème juridique soulevé par nos collègues du groupe Les Républicains. Le Sénat a intérêt à statuer sur cet aspect particulier de la responsabilité du fait des choses, quitte à ce que ce travail soit un jour intégré à une réforme plus vaste de la responsabilité civile. En commission, notre rapporteur nous a proposé d'intégrer le nouveau dispositif prévu dans la proposition de loi non pas dans le code de l'environnement, mais dans le code du sport. Nous souscrivons à cette modification, d'autant plus que ce code prévoit déjà, dans son article L. 321-1-3, une exonération, pour les pratiquants d'une activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels à l'encontre d'autres pratiquants du fait des choses sous leur garde. Rappelons au passage que cette évolution de 2012 était, elle aussi, issue d'une initiative parlementaire. Sur le plan juridique, l'évolution de la matière qui nous occupe aujourd'hui a été largement bouleversée par un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en 2010 et réduisant le champ d'application de la théorie des risques acceptés. Depuis ce revirement, la responsabilité du fait des choses a désormais vocation à s'appliquer à l'ensemble des dommages causés par le fait d'une chose, quelle que soit la nature de celle-ci, quel que soit le dommage causé et quelle que soit l'activité qui en a été l'occasion. Les effets de cette décision se sont rapidement fait sentir avec une forte augmentation des primes d'assurance de certaines fédérations, notamment en matière de sport mécanique. Force est de constater que la problématique que nous examinons ce soir est très spécifique, puisque les « choses » dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas des matériels de sport : il ne s'agit pas de la responsabilité des dommages causés par une raquette de tennis ou une moto de compétition ... Ces hypothèses, plus classiques, ont déjà donné lieu à de très nombreuses décisions judiciaires. Ici, il est en fait question, au travers de la notion juridique de « chose », d'éléments qui composent l'environnement naturel d'une pratique sportive, en l'occurrence un rocher sur une paroi d'escalade. On comprend bien que le débat n'est pas tout à fait de même nature. On comprend surtout qu'en désignant comme juridiquement responsable une fédération sportive pour des dommages qu'elle ne pouvait ni prévoir ni éviter, on la place dans une situation intenable. L'objectif de cette proposition de loi est très simple, mes chers collègues : trouver le bon aménagement juridique permettant de sauvegarder et de permettre le développement d'activités sportives et de nature. Vous avez ainsi évoqué, madame la secrétaire d'État, le nombre de pratiquants dans notre pays de ce type d'activités. Je tiens à remercier notre rapporteur de la qualité de son travail, la finesse de son analyse juridique et l'intelligence des apports faits à la proposition de loi initiale. Il nous propose aujourd'hui un dispositif qui pourra sans doute encore être amélioré de la navette parlementaire, mais qui lance le débat et souligne l'implication du Sénat sur cette problématique très importante pour le développement économique et touristique de nos territoires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer en commission, j'aime les premiers de cordée. Non pas dans l'acception macroniste de la formule, ... Cela viendra ! ... mais au sens littéral du terme. Je suis moi-même grimpeur, mais comme cela n'emporte pas d'obligation de déport ou de conflit d'intérêts, je poursuis mon propos. Pour poser les termes du débat qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai choisi de partir du nom qu'on donne en escalade à celui qui se trouve à l'autre bout de la corde, tout en bas : il s'agit de l'assureur. l'assureur. Ce terme résume à lui seul toutes les interrogations auxquelles cette proposition de loi veut apporter des réponses, soit la prise de risque, la responsabilité qui y est liée et le financement des dommages en cas d'accident. Autrement dit, qui pratique, qui sécurise et qui paye ? Ce texte trouve notamment son origine dans un accident d'escalade à Vingrau et dans une décision de justice s'y rapportant. Mais les questions posées intéressent tous les pratiquants de sport de pleine nature, l'ensemble des fédérations qui en régissent la pratique, les propriétaires de sites naturels et les collectivités territoriales qui en assurent le développement et la promotion. Plusieurs questions philosophiques sous-tendent nos débats aujourd'hui. Quelle place accordons-nous à la prise de risque dans notre société, notamment dans les espaces naturels ? Quelle part d'acceptation du risque de la part des pratiquants eux-mêmes ? Sur ces sujets, qu'est-ce qui doit relever de la responsabilité individuelle ou de l'assurance d'un tiers ? Jusqu'où les fédérations et les collectivités doivent-elles être responsables des pratiques individuelles ? Quel est le juste coût des assurances que doivent prendre en charge les pratiquants ? La première des questions que nous nous sommes posées en commission était : devons-nous légiférer sur la base d'un cas précis et d'une décision de justice, toujours en appel ? Autrement dit, faut-il attendre la Chancellerie et la prochaine réforme du droit de la responsabilité ? Nous avons

Pourtant, les textes de 1804, comme la construction jurisprudentielle qui les accompagne, ne sont plus à même de répondre à la complexité des situations auxquelles nous devons faire face aujourd'hui. Vous avez sans doute lu le récit dans la presse cette semaine du sauvetage héroïque d'Élisabeth Revol. Son histoire a bien commencé, quand elle est devenue la première femme à réussir l'ascension hivernale du Nanga Parbat, en compagnie d'un alpiniste polonais.

Elle a été rejointe par d'autres ressortissants polonais venus à sa rescousse de nuit, à la lampe frontale, dans des conditions dantesques. Cette histoire, terrible, ne nous intéresse pas aujourd'hui que par son contexte : les montagnes françaises ne sont pas l'Himalaya et l'initiative législative du jour n'aurait que peu d'impact au Pakistan. Pakistan. Elle nous interpelle par les messages qu'elle porte. Nul n'imaginait qu'une opération de sauvetage dans l'Himalaya puisse être payée grâce à un appel au financement participatif, à hauteur de 50 000 dollars, en temps réel, au moment même du drame vécu par Élisabeth Revol sur le Nanga Parbat. Les pratiques sportives actuelles, dans l'environnement juridique contemporain, requièrent des réponses nouvelles. J'ai le sentiment que cette proposition de loi nous les apporte. Je crois également que le travail de précision juridique, apporté avec beaucoup de minutie par notre rapporteur, va dans le bon sens. Le grand grimpeur et alpiniste italien Reinhold Messner nous dit que « la montagne n'est ni juste, ni injuste, elle est dangereuse Sur la question du risque lié à la pratique des sports de pleine nature, nos efforts doivent précisément porter sur la juste responsabilité de chacun des acteurs concernés. Cela vaut pour les risques ordinaires comme pour les risques exceptionnels. Pour la clarté de la démonstration, je veux dresser le tableau noir, dans le champ de l'escalade, des conséquences possibles d'une situation où le régime de la responsabilité sans faute continuerait à prévaloir une fédération, la Fédération française de la montagne et de l'escalade, qui suspend tout ou partie des 800 conventionnements qui la lient à des propriétaires partout en France ; des propriétaires qui interdisent l'accès à leurs sites un niveau d'équipement et de sécurisation des sites qui diminue ; des pratiques sauvages ou clandestines qui prospèrent ; des collectivités

Au-delà des risques en matière d'accidentologie, ou des crispations possibles entre propriétaires et pratiquants, il faut considérer sérieusement cette perte de ressource réelle de développement local pour des communes, intercommunalités ou départements qui auraient été prêts, littéralement, à « investir dans la pierre Vous aurez compris que je prône au nom de mon groupe- c'est de circonstance s'agissant d'escalade -une position équilibrée. Le texte que nous étudions interroge à ce titre, en premier et en dernier lieu, les pratiquants. L'escalade, la randonnée et le VTT font partie des rares pratiques totalement libres d'accès et gratuites. C'est une chance et un rare privilège dans un monde de plus en plus marchand et je suis, comme beaucoup d'autres, très attaché à ces deux caractéristiques. On peut considérer à l'échelle nationale que la moitié de la population française pratique la marche ou la randonnée. Trois Français de plus de quinze ans sur quatre déclarent, en 2016, pratiquer un sport de nature, soit 34,5 millions de personnes. La contrepartie de ce libre accès et de cette gratuité doit sans doute être recherchée dans l'acceptation sociale d'un risque raisonnable. Cela renvoie à la nécessité, dans le cadre de pratiques non encadrées, d'avoir des pratiquants conscients, formés, assurés. Dans le modèle qui nous intéresse, le rôle des fédérations est central sur ces trois points. Car des pratiquants mieux formés, davantage responsabilisés, cela signifie moins de risque d'accident. Vous aurez donc compris que tout le monde est concerné par ce texte : l'alpiniste chevronné, le randonneur occasionnel, le « VTTiste » du dimanche. Je souhaite que l'on puisse continuer à emprunter un sentier de grande randonnée, pour aller à Compostelle ou ailleurs, sans devoir se détourner d'un chemin qu'un propriétaire inquiet aurait interdit d'emprunter et que l'on puisse initier des enfants à l'escalade sans analyse juridique préalable. Au nom de mon groupe, j'apporte mon soutien à cette proposition de loi de M. Retailleau, ... Très bien ! ... le président d'un groupe avec lequel je suis souvent en désaccord, mais avec lequel il m'arrive aussi de tomber d'accord sur des sujets de niche, comme cette proposition de loi ou l'importance du jeu vidéo Les amendements adoptés en commission me satisfont. Le rapporteur a fait le choix de définir la notion de faute dans un sens plus restrictif qu'initialement prévu, ce qui semble adapté à l'activité visée. En ce qui concerne l'articulation avec l'actuel article L. 365-1 du code de l'environnement, on comprend que la cohabitation de deux dispositifs risquerait de créer des règles contradictoires.

aux assureurs, aux randonneurs et à tous ceux qui font des espaces naturels leur terrain de jeu privilégié.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est avec une certaine perplexité que j'aborde cette

forte artificialisation d'un certain nombre de ces espaces qui amoindrit les espaces de nature. Nous assistons à des demandes de plus en plus nombreuses de manifestations sportives, souvent axées sur la performance. En même temps, nous constatons un grand attachement de nos concitoyens à la nature et aux espaces naturels. On a déjà aussi évoqué l'intérêt touristique pour l'attractivité des territoires de ces espaces naturels.

générale de la société. Dès que l'on reçoit un gravier sur le coin de la tête, on se demande comment faire réparer le préjudice de cette atteinte à son intégrité physique ... Les contentieux en responsabilité exposent les propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels, malgré toute l'information fournie et les précautions prises. Si cette tendance se confirmait, certains propriétaires ou gestionnaires d'espaces naturels

le choix fait par la commission des lois, que je peux comprendre et qui a une pertinence juridique indiscutable, me paraît, et je

par les promeneurs, les sportifs, et de favoriser également la sécurité des gardiens de ces sites, qui ne pouvaient pas voir leur responsabilité engagée à tout propos dès lors qu'ils ouvraient très largement ces espaces

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir nous place devant la question de la prise en charge des risques individuels par la société, sous l'angle spécifique de la pratique des sports de nature. De nos jours, ces activités progressent en nombre et rassemblent beaucoup d'adeptes, y compris sur ces travées. À titre d'exemple, la Fédération française de randonnée pédestre compte 242 000 adhérents et la Fédération française de la montagne et de l'escalade quelque 96 000. Plus de trois Français sur quatre de plus de quinze ans déclarent pratiquer régulièrement une activité de pleine nature. Les auteurs de la proposition de loi l'ont souligné, il s'agit également d'un facteur majeur d'attractivité, encouragé par la loi, pour bon nombre de nos territoires. nos territoires. Sur les territoires de montagne en particulier, la loi du 9 janvier 1985 permet de limiter le droit de propriété au nom de l'activité sportive, l'objectif étant de favoriser le développement du tourisme. Cependant, le développement de ces activités n'est pas sans causer certaines difficultés. En premier lieu, et c'est l'objet de cette proposition de loi, il existe une difficulté juridique liée à la mise en cause de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels en cas d'accidents. La pluralité des situations juridiques s'appliquant à la pratique des sports de nature ne facilite pas l'analyse, selon qu'il s'agisse de pratiques encadrées par une association ou une entreprise ou d'une pratique « sauvage » et selon l'état des relations entre le propriétaire du site naturel, public ou privé, et son gestionnaire. Lorsque ces activités sont dangereuses, elles devraient faire l'objet d'un encadrement minimal, ce qui n'est d'ailleurs pas contraire à l'objectif de dynamiser le tissu économique rural. les activités sportives « sauvages » pratiquées hors des périmètres balisés par le propriétaire ou le gestionnaire des sites régulièrement désigné par le propriétaire devraient plutôt engager la responsabilité des sportifs concernés. Si je prends l'exemple du département que je connais le mieux, celui du Puy-de-Dôme, où les volcans de la chaîne des Puys sont dans leur quasi-totalité des espaces privés, comment des propriétaires pourraient-ils courir un risque juridique démesuré alors qu'ils offrent leurs parcelles aux activités de nature, sans que la fréquentation soit réellement maîtrisable ? L'engouement pour les sports de nature accroît considérablement la pression sur eux qui, dans nombre de cas, n'ont parfois pas consenti à y accueillir du public. Le régime actuel de responsabilité sans faute pourrait, en outre, se révéler très coûteux pour les gardiens de sites naturels, comme dans le cas de l'exemple retenu par Bruno Retailleau et ses collègues, si leur responsabilité devait être systématiquement recherchée devant les tribunaux après chaque accident. C'est pourquoi il est utile aujourd'hui de s'interroger sur une évolution du régime de responsabilité. Comme l'ont déjà souligné certains membres de la commission des lois, il s'agit d'ailleurs plus d'une conséquence de l'aversion au risque de notre société et de logiques assurantielles sous-jacentes que de la volonté des pratiquants de ces sports extrêmes, familiers de la prise de risque. Il est donc nécessaire de parvenir à une rédaction équilibrée, qui ne limite pas la pratique des sports de nature, pas plus qu'elle ne déresponsabilise les propriétaires ou gestionnaires de sites naturels, ni les pratiquants de telles activités sportives. Utiliser un espace à à des fins de loisirs est un droit qui doit s'accompagner de devoirs, le premier étant de respecter la propriété d'autrui, en étant responsable de ses actes et en faisant preuve de prudence. De ce point de vue, la rédaction proposée par le Gouvernement offre un bon compromis, que nous soutiendrons. En second lieu, cette discussion ne doit pas occulter une autre responsabilité collective liée à la pratique des sports de nature et des activités de plein air. L'adaptation du droit de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites ouverts au public ne doit pas s'appréhender aux dépens de la nécessaire préservation de ces espaces, déjà fragiles par nature et parfois mis à rude épreuve par les pratiques sportives. Sur ce sujet, la responsabilité des gestionnaires de sites ne doit pas être totalement exonérée. Il y va de la pérennité de ces espaces et de notre capacité à les transmettre aux générations futures. Un meilleur partage des responsabilités doit être trouvé. Enfin, un partenariat avec les propriétaires est nécessaire pour permettre une meilleure signalétique et une meilleure information des usagers. Le soutien à l'attractivité des territoires et au développement de cette économie touristique passe par l'accompagnement des gardiens de sites naturels.

nous nous apprêtons à examiner une proposition de loi émanant du président Bruno Retailleau et de ses collègues et visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Aujourd'hui, les propriétaires fonciers qui laissent libre accès à leur domaine, sans toutefois l'autoriser, peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle dans les conditions de droit commun, dans l'hypothèse où des sportifs ou des promeneurs viendraient à se blesser sur leur terrain. Leur responsabilité peut ainsi être recherchée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, relatif au régime de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Il résulte, à ce titre, d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le gardien est celui qui en a l'usage, le contrôle et la direction au moment du fait dommageable, et que le propriétaire est présumé gardien. La seule manière alors pour ce dernier de s'exonérer totalement de sa responsabilité est de prouver un cas de force majeure, ou, à tout le moins, de s'en exonérer partiellement en démontrant que la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Il existe actuellement une exception à ce principe général de responsabilité civile à l'article L. 365-1 du code de l'environnement, lequel prévoit un régime dérogatoire de responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de certains types d'espaces, tels que les parcs nationaux ou les réserves naturelles. Rappelons pour mémoire qu'un article L. 160-7 alinéa 4 du code de l'urbanisme, abrogé depuis lors par une ordonnance du 23 octobre 2015, prévoyait que la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes de passage des piétons sur le littoral, définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du même code, ne pouvait être engagée au titre des dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. En tout état de cause, cet aménagement de la responsabilité des propriétaires étant limité, il est actuellement recommandé aux propriétaires de souscrire une assurance de responsabilité civile pour leur éviter de supporter les conséquences dommageables en cas de préjudice. Poursuivant un objectif louable, celui de favoriser le développement des sports et activités de nature qui représentent un attrait touristique majeur pour de nombreuses collectivités territoriales, la proposition de loi prévoyait initialement dans un article unique d'étendre l'exception prévue à l'article L. 365-1 du code de l'environnement aux propriétaires et gestionnaires de sites naturels pour les dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisir ou de sports de nature. La commission des lois a souhaité retenir une autre rédaction et exclure la mise en cause au titre de leur responsabilité sans faute, fondée sur le premier alinéa de l'actuel article 1242 du code civil, de ces propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public et dans lesquels s'exercent les sports de nature ou les activités de loisir, en cas de dommages subis par leurs pratiquants. La commission a préféré l'application du régime de la responsabilité pour faute. Il a également été décidé d'introduire ce dispositif dans le code du sport. Si le groupe La République En Marche reconnaît l'intérêt évident d'une telle proposition, nous pensons néanmoins que son insertion dans un processus plus global de réforme de l'ensemble des règles régissant la responsabilité civile, portée prochainement par Mme la garde des sceaux, aurait plus de sens. Aussi, et parce que vous le reconnaissez vous-même monsieur le rapporteur, ce contentieux est peu abondant, en attendant le jugement en appel, voire en cassation, du cas d'espèce ayant motivé la proposition de loi, nous choisissons de réserver notre position.

la question soulevée ce soir n'est pas nouvelle. Le régime de responsabilité des propriétaires de sites naturels avait déjà été débattu en 1984 lors de la discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en 2005 dans le cadre du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux et, plus récemment en 2006, lors de l'examen du projet de loi relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. Toutefois, cette proposition de loi a le mérite d'aborder le paradoxe entre la demande croissante d'accès à des sites naturels préservés d'un point de vue écologique et paysager, et une moindre acceptation, supposée, des risques que cela comporte.

Or le propriétaire ou le gestionnaire d'un site naturel ouvert au public peut être reconnu responsable, sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, si un dommage est causé lors de la circulation du public sur sa propriété, qu'il l'ait ou non autorisée, s'il n'a pas explicitement défendu l'accès à son terrain. Cette responsabilité de l'article 1242, alinéa 1, du code civil est une responsabilité sans faute, dite « responsabilité objective ». Du seul fait de son caractère de gardien de la chose, le propriétaire pourra être reconnu responsable d'un dommage. C'est sur le fondement de cet article, dans un jugement datant de 2016, que le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la Fédération française de la montagne et de l'escalade entièrement responsable d'un accident grave causé par la chute d'un bloc rocheux sur un site naturel d'escalade survenu en 2010 et l'a condamnée solidairement avec la compagnie d'assurance à verser aux victimes une somme de 1,2 million d'euros à titre de dommages et intérêts. Cette jurisprudence a suscité un émoi certain dans mon département. Si elle devait être confirmée, elle porterait en germe le risque d'une interdiction d'accès à de nombreux sites naturels. C'est pourquoi il nous est proposé de préserver l'accès à ces sites naturels au travers d'une modification, un allégement du régime de responsabilité que peuvent encourir leurs propriétaires ou gestionnaires. Si nous partageons les craintes du rapporteur, il faut noter que cette jurisprudence n'est pas stabilisée, puisqu'il s'agit d'un jugement de première instance. D'ailleurs, le 2 février 2017, dans une autre affaire où la responsabilité de l'Office national des forêts était recherchée sur le même fondement de la responsabilité sans faute, à la suite d'un accident dont fut victime un adolescent alors qu'il pratiquait le VTT sur un circuit « sauvage » dans une forêt domaniale, la cour d'appel de Versailles a, au contraire, confirmé le jugement en première instance déboutant la victime et ses parents. Dès lors, l'examen de cette proposition de loi peut sembler prématuré, car il y a très peu de contentieux et de condamnations sur le fondement de l'article 1242. En outre, cet article n'implique pas une responsabilité automatique du propriétaire ou du gestionnaire, car le juge va se livrer à un examen approfondi des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, pour décider si le propriétaire est ou non civilement responsable. Ainsi, si elle semble extrêmement extensive, la responsabilité du fait des choses est toutefois encadrée par le juge, comme le souligne un rapport un groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur la responsabilité civile : « Les juridictions ne font pas un usage abusif de la responsabilité du fait des choses, qui reste encadrée par certains garde-fous. De plus, nous ne pouvons éluder la question de l'opportunité de légiférer pour infléchir un jugement de première instance, qui n'est donc pas définitif. Certes, le rapporteur précise qu'il s'agit d'anticiper de futurs problèmes. Toutefois, cela peut sembler peut sembler précipité, car lorsque le législateur intervient pour remettre en cause une politique jurisprudentielle, il s'agit généralement d'une jurisprudence confirmée en cassation. Enfin, il est très difficile d'appréhender la réaction des assureurs face à une responsabilité fondée sur la faute. À l'opposé de l'objectif, ne risque-t-on pas de voir se multiplier des mouvements de sécurisation des sites naturels pour éviter une telle responsabilité ? De même, pour reprendre les mots de chercheurs sur la question, « la notion de faute est par ailleurs évolutive dans le temps et l'espace : elle ne peut ainsi être engoncée dans un texte trop précis, sa silhouette se dessinant au gré des décisions de justice et des évolutions sociétales ». Ainsi, de nombreuses interrogations demeurent même après le passage en commission. Toutefois, la question de la confiance des propriétaires et de l'accès aux sites naturels est une véritable problématique des zones de montagne et la crainte des propriétaires et des gestionnaires après la condamnation de la FFME en première instance est réelle et peut renforcer les difficultés déjà existantes d'accès aux sites naturels privés. Pour ces raisons, l'amendement du Gouvernement nous paraît un bon compromis. Cependant, dans l'intérêt général, et malgré ces nombreuses interrogations, nous voterons cette proposition de loi réécrite par la commission.

Je soutiens bien sûr la présente proposition de loi, déposée par mes collègues Bruno Retailleau et Michel Savin, visant à adapter le droit de responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Nous n'avons effectivement pas besoin d'attendre la réforme de la responsabilité civile annoncée par le Gouvernement pour lancer la réflexion sur la responsabilité du fait des choses. Cette proposition de loi est une occasion pour le Sénat de se saisir de la question. En effet, il n'est pas normal que les propriétaires ou gestionnaires de ces terrains engagent leur responsabilité sans faute pour des faits qui ne relèvent pas de leur volonté, sachant de surcroît qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler efficacement les accès et les activités s'y déroulant, coupables de n'avoir pas pu prévoir les aléas de la nature. de la nature. Cela peut conduire au jugement que vous connaissez et sur lequel je ne m'attarderai pas, lorsque le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné le 14 avril 2016, la Fédération de la montagne et de l'escalade, gestionnaire d'un site naturel pour le compte d'une commune, à indemniser à hauteur d'un million d'euros la victime malheureuse d'un accident d'escalade causé par le détachement d'un bloc de pierre de la paroi sur laquelle il progressait. Les sites naturels ouverts au public devraient pouvoir continuer de l'être sans faire peser une épée de Damoclès d'ordre juridique et financier sur la tête de ceux qui en sont les gardiens. Il faut renouer avec la vision selon laquelle, dans le monde du sport et, en particulier, du sport de nature, le devoir de protection porte sur les risques créés par autrui, non sur ceux qui sont liés aux activités auxquelles l'individu participerait volontairement. Quand on pratique ce genre de sports ou de loisirs, on est conscient que l'environnement dans lequel on évolue est périlleux. Un simple promeneur est d'ailleurs lui aussi vigilant quand il s'aventure sur ces sites naturels. Si vous choisissez de marcher en forêt, vous savez pertinemment que vous devrez regarder où vous mettez les pieds. Comme le rappelait en commission, notre collègue Jérôme Durain, même Reinhold Messner, premier alpiniste à avoir gravi les quatorze sommets culminant à plus de 8 000 mètres d'altitude, disait que « la montagne n'est ni juste ni injuste, elle est dangereuse Une dérive de la législation actuelle est la déresponsabilisation des usagers. Si dans l'esprit de tous un randonneur venait à devenir un simple consommateur de sport sur un terrain qui lui serait en quelque sorte mis à disposition, comme un tennisman pourrait se plaindre du mauvais état du cours pour lequel il paie, il ne prendrait alors plus en considération les possibles risques liés à l'environnement naturel dans lequel il se trouve, s'attendant à ce que tout soit entièrement organisé. Ayant l'habitude d'être « surencadré » dans un terrain naturel aménagé dans lequel il se comporte comme un consommateur, il peut être tenté de manière tout à fait inconsciente d'avoir la même attitude en s'aventurant dans les espaces naturels non aménagés. Combien de skieurs se mettent-ils en danger chaque année en hors-piste ? Par conséquent, la lourde responsabilité sans faute des propriétaires et gestionnaires les incite à entreprendre un aménagement excessif visant à sécuriser les sites et ayant pour conséquence une dénaturation regrettable de ceux qui sont censés rester des espaces naturels. Il y va de l'avenir de nos beaux paysages français. Nul besoin d'aller loin de Paris, imaginez-vous la forêt de Fontainebleau défigurée par une série de filets, de barrières, de rambardes et de signalisations de couleur en tous genres D'autres, au contraire, préfèrent tout simplement fermer l'accès de ces sites au public, freinant ainsi le développement des sports de nature et des activités de loisirs en plein air en évolution perpétuelle, alors que notre immense patrimoine naturel nous offre tant de possibilités.

constituent un atout touristique majeur, comme dans beaucoup de collectivités territoriales. Le temps libre s'accroît, les techniques et le matériel progressent, les connaissances se diffusent et, par conséquent, le niveau de pratique augmente. Il est de notre devoir de protéger ces sites encore ouverts au public, leurs propriétaires, leurs gestionnaires, les activités de sports et de loisirs qui y sont proposées, les emplois qui y sont associés et la dynamique touristique qui y est liée. C'est pourquoi il semble nécessaire d'apporter au plus vite une solution à la faiblesse du dispositif légal actuel. Je voterai donc en faveur de la présente proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Très bien

Il vise à réintroduire cette disposition dans ledit code, tout en répondant aux inquiétudes exprimées par le rapporteur, lors de la réunion de la commission des lois, quant au caractère trop vague

instaurant une disposition excluant la mise en cause des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité sans faute pour des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation du public ou de la pratique d'activités de loisirs ou de sports de nature, tout en respectant le choix de la commission des lois d'introduire une disposition identique à l'article L. 311-1

d'abord rendre hommage à Jérôme Bignon, pour sa volonté de trouver une solution à une situation qui, il le rappelait tout à l'heure dans la discussion générale, est complexe.

Le troisième alinéa de cet amendement vise à dupliquer cette rédaction, en remplaçant les termes « sites naturels » par les termes « espaces naturels ouverts au public

le texte de l'actuel article L. 365-1 du code de l'environnement, mais seulement pour la responsabilité administrative. Cette disposition invite ainsi le juge administratif à prendre en compte les particularités des espaces naturels énumérés

le législateur n'a pas besoin de l'inviter à le faire ... Par ailleurs, ce troisième alinéa n'est pas adapté à la responsabilité administrative, qui obéit à des règles particulières.

Cette fois, le dispositif de responsabilité pour faute, introduit au début de l'article L. 365-1, concernerait, de manière générale, non seulement les espaces naturels ouverts au public, mais encore une liste de sites particuliers, énumérés pour la plupart dans l'actuel article L. 365-1 du code de l'environnement. Cette rédaction pose plusieurs difficultés. En premier lieu, les deux alinéas du dispositif proposé s'articulent mal entre eux ; ils répètent la même chose, avec des termes un peu différents, ce qui rend le dispositif peu compréhensible. Ils me semblent donc contraires aux objectifs de clarté et d'intelligibilité de la loi. En second lieu, cette rédaction, par l'imprécision des termes utilisés, encourt les mêmes critiques que celles qui ont été formulées à l'encontre de la proposition de loi dans sa rédaction initiale. Par ailleurs, cette rédaction va bien plus loin que l'objectif des auteurs de la proposition de loi- favoriser le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air qui se déroulent dans le domaine privé des personnes publiques ou privées -, puisqu'elle pose un principe général d'exonération de responsabilité civile et administrative

sur le fond, les dispositions proposées excluent involontairement l'application du régime de responsabilité du fait des choses, même pour les simples promeneurs.

par le fait que ces nouvelles dispositions auraient vocation à coexister avec le nouvel article introduit par la présente proposition de loi dans le code du sport. Aussi, dans ce contexte et eu égard aux changements à venir sur le droit de la responsabilité civile,

sans préjudice d'une modification ultérieure du régime de responsabilité spécifique applicable aux activités sportives, l'article L. 365-1 du code de l'environnement pourrait donc être, selon nous, maintenu. Néanmoins, au regard des préoccupations exprimées,

plus large, d'espace naturel. Enfin, cette nouvelle rédaction prendrait en compte les espaces restés vierges de tout aménagement dans un objectif de préservation du caractère naturel de l'espace. En effet, la disposition existante ne concerne expressément que les espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements, ce qui peut susciter des difficultés d'interprétation.

pour rappel, que cet article invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels. Selon cet article, cette responsabilité doit être appréciée « être appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique ». Ce dispositif a une portée normative limitée, puisqu'il pointe seulement les éléments factuels que le juge doit prendre en considération pour se prononcer. Or c'est bien le rôle du juge que d'apprécier, pour chaque contentieux, les circonstances de l'espèce. Le législateur n'a, je le de l'inviter à le faire. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité aller plus loin que cette hypothèse-là, et aller jusqu'au remplacement de la responsabilité du fait des choses par la responsabilité pour faute. Cet amendement ne permet pas d'atteindre l'objectif des auteurs de la proposition de loi et de la commission des lois,

une solution sage, qui permettrait de ne pas se précipiter. Rappelons-le, l'affaire qui a en partie motivé la proposition de loi que nous examinons